Il aura suffi de quelques semaines et d’un dumping extrême des fabricants chinois de panneaux photovoltaïques pour détruire son modèle économique, pourtant solide. Face à cette situation, l’État reste muet.

voir le jour que si l’Europe se met vraiment en ordre de bataille en matière douanière contre le dumping chinois, ce qui est très loin d’être acquis. En attendant, les entreprises les plus innovantes meurent, faute de soutien.

Nous savons que la transition territoriale est au cœur de la planification écologique : le ministre Christophe Béchu le martèle lors de toutes les COP régionales. Nous l’avions d’ailleurs souligné au moment de l’examen

deux questions précises. Les décrets sur le partage de la valeur vont ils être publiés ? Allez vous préserver la filière photovoltaïque française existante ? Il y a urgence climatique ! Or, d’après le Haut Conseil pour le climat (HCC), vous seriez en train de l’oublier.

La classe politique, dans son ensemble, a exprimé sa profonde indignation et sa compassion après la mort de Shemseddine le vendredi 5 avril, à Viry Châtillon, dans mon département de l’Essonne. La disparition tragique de cet adolescent de 15 ans, sauvagement massacré par cinq individus, dont quatre mineurs, vient malheureusement s’ajouter à une liste déjà trop longue et insupportable. Au delà des éternelles déclarations médiatiques, d’une fermeté de façade qui ne trompe plus personne, du gigantesque déni idéologique qui paralyse l’action publique, publique, des sempiternelles déclarations solennelles du Président de la République jurant que « la main de l’État ne tremblera pas » et que « l’école doit rester un sanctuaire », alors qu’elle est devenue un coupe gorge

de nos personnels, sont arc boutés précisément pour que l’école reste un lieu de sécurité et de sérénité. C’est en tout cas la volonté du Gouvernement, et nous nous employons à faire en sorte qu’il en soit ainsi. que vous avez soulignée, des instants qui nous ont réunis auprès de Shemseddine lorsque nous nous sommes rendus à Viry Châtillon. J’étais présente au moment où la mort de cet élève a été annoncée à ses camarades. J’ai pu, aux côtés de la communauté éducative, partager leur douleur et dire l’infinie tristesse qui a saisi le collège. Monsieur le sénateur, ce ne sont pas que des mots ! Lorsque l’on appartient à une famille, on vibre de ces sentiments

un bouclier fondé sur les forces de l’ordre, le travail pédagogique, le respect des valeurs républicaines et l’ensemble des dispositifs de formation, de prévention, de protection juridique

Les plus grands spécialistes ont posé les diagnostics depuis bien longtemps ! L’ultraviolence juvénile n’est pas le fruit du hasard. Partout, l’autorité est bafouée et l’anomie nous guette. Alors, au moment même où les piliers de notre société sont consciencieusement dynamités les uns après les autres, l’heure n’est plus aux missions flash ou à je ne sais quel autre sabir ! L’urgence commande désormais d’agir. Mais quand allez vous enfin ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans notre pays ?

Ces scénarios illustrent les possibles conséquences de l’inaction face aux effets du changement climatique, qui obligeront nombre de nos compatriotes de l’Hexagone comme des outre mer à changer de logement ou à l’adapter. Parmi les personnes les plus affectées figurent les habitants de mon département, la Guadeloupe, où 500 foyers, composés majoritairement de personnes âgées, voient leur vie menacée du fait de leur exposition aux phénomènes climatiques naturels.

bail concerne avant tout les propriétaires. Or la majorité des victimes de l’érosion en Guadeloupe ne le sont pas ; elles ne peuvent donc pas bénéficier de ce dispositif de droit commun. Monsieur le ministre, face à l’ampleur de ces scénarios, l’anticipation s’impose. Les acteurs locaux sont déjà prêts et engagés, mais ils ont besoin de ressources. Quelles sont les mesures prévues pour les accompagner et rendre le relogement de ces familles le moins pénible possible ? Quelles actions l’État mettra t il en place pour mieux appréhender ce phénomène et renforcer l’information des acquéreurs

La parole est à Mme Laure Darcos, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. Ma question s’adresse à Mme la ministre de l’éducation nationale Madame la ministre, Shemseddine avait 15 ans. Il sortait de son cours de musique quand il a été tabassé à mort par plusieurs jeunes encapuchonnés pour la simple raison qu’il fréquentait une jeune fille et que cela déplaisait aux frères Présente, comme vous, vendredi sur les lieux de ce meurtre barbare aux côtés de mon ami Jean Marie Vilain, maire de Viry Châtillon, j’ai croisé à la sortie du collège ses camarades, en pleurs, incrédules et terrorisés. Malgré leur désarroi, ils posaient tous la même question : « À qui le tour ? Au cœur d’une société déboussolée, l’école a vocation à être un sanctuaire de la République, formant génération après génération nos enfants au respect mutuel et aux droits humains élémentaires, où les élèves comme leurs professeurs se sentiraient en sécurité. Les communes ne cessent d’investir dans les quartiers populaires pour que chacun, dans sa différence, vive en harmonie avec les autres. L’effort consenti est colossal. Je peux témoigner que le maire de Viry Châtillon et son équipe développent de nombreuses actions dans leur ville pour que les habitants s’y sentent heureux. Alors, que Alors, que faire de plus ? Que faire de mieux ? Comme vous tous ici, je me sens découragée devant l’ultraviolence de mineurs de plus en plus jeunes. Ceux ci perdent le sens du bien et du mal, notamment à travers les réseaux sociaux, qui influencent leurs comportements et répandent de manière virale des rumeurs abjectes sur leurs camarades. Pouvons nous accepter de cette jeunesse une haine des forces de police, des pompiers, des élus et de leurs enseignants ? Pouvons nous nous habituer à cet ensauvagement, qui vire à la barbarie ordinaire ? Bien sûr, il faudra punir ces assassins très sévèrement et, autour d’eux, rappeler qu’en France il existe un devoir fondamental de respect de la vie d’autrui. Par ailleurs, en 2024, l’infantilisation des femmes par un patriarcat moyenâgeux n’a pas sa place dans la République, et l’éducation à la sexualité à l’école doit pouvoir être enseignée en toute sérénité. Notre indignation ne ramènera pas Shemseddine à la vie. Sa maman, une veuve courageuse, son frère et sa sœur sont brisés à tout jamais. Pouvons nous espérer que ce drame serve à une véritable prise de conscience et à un sursaut collectif ?

en ligne. Basées à l’étranger, ces entreprises profitent de l’absence de régulation française pour cibler un jeune public et réaliser des profits importants. L’absence de règles applicables à ces jeux de casino en ligne surexpose nos concitoyens à la captation de leurs données personnelles, à la fraude aux moyens de paiement, à l’installation de programmes informatiques malveillants, au non paiement des gains et, au travers de la cybercriminalité, participe au financement d’activités terroristes. Ces sites frauduleux posent également de sérieux problèmes en termes de santé publique : près de 80 % de leurs bénéfices sont réalisés grâce à des joueurs ayant une pratique de jeu à risque ; un quart d’entre eux sont âgés de 18 à 24 ans.

efficace d’assécher l’offre illégale. L’exemple des Pays Bas montre que 85 % de ces sites ont disparu après cette légalisation et que celle ci n’a absolument pas fragilisé les casinos physiques, bien au contraire.

il faut le dire de manière très claire, l’eau est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Les agences régionales de santé (ARS) assurent chaque jour des dizaines et des dizaines de contrôles sanitaires sur l’ensemble du territoire. Votre question fait référence à la conformité sanitaire de l’eau en bouteille produite par le groupe Nestlé Waters. Des révélations récentes ont mis en évidence que cette société aurait eu recours à des traitements de l’eau interdits par la réglementation. Une enquête préliminaire pour tromperie a été ouverte à l’encontre de cette entreprise par le parquet d’Épinal. Bien évidemment, je ne commenterai pas ici une affaire judiciaire en cours. Toutefois, je veux redire que les contrôles sanitaires réalisés par les ARS sur les deux sites qui auraient utilisé des traitements interdits ont toujours témoigné de la conformité sanitaire de l’eau embouteillée. Je tiens donc à rassurer nos concitoyens les eaux mises en vente respectaient, et respectent, les normes sanitaires. La question est seulement de savoir si elles respectent les normes applicables aux eaux de source ou aux eaux minérales ; la justice est saisie

À cet effet, une note d’appui scientifique et technique a été produite par l’Anses, afin d’aider les ARS à définir les paramètres et les conditions de cette surveillance renforcée de la sécurité sanitaire des filières d’eau conditionnée. Ce plan est actuellement mis en œuvre à la demande des ARS, et cela sur les deux sites.

dans une tribune signée conjointement avec le président égyptien al Sissi et le roi Abdallah de Jordanie, le Président de la République vient d’appeler à un cessez le feu à Gaza et à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. demande l’arrêt du processus de colonisation et affirme sa volonté de faire aboutir une solution à deux États. Cette prise de position n’est pas anodine. Elle tient compte de l’exigence mondiale d’un arrêt de la guerre et des massacres en cours à Gaza où, il faut le rappeler, plus d’enfants ont été tués en quatre mois qu’en quatre ans de conflits à travers le monde. Mais après ? Aussi fortes soient elles, les déclarations restent sans portée si les décisions ne suivent pas. Depuis six mois, aucune déclaration, aucune résolution de l’ONU, aucune injonction de la Cour internationale de justice, aucune négociation, y compris celle qui a lieu au Caire en ce moment, n’ont fait

Il faut joindre les actes aux paroles et aux écrits. Aussi, je vous le demande, monsieur le ministre : agissez concrètement et fermement. Faites immédiatement pression pour qu’Israël applique les mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice

Que compte faire le Gouvernement, au delà des 4 100 nouvelles places créées sur les 15 000 places prévues en 2017 ?

nouvelles places de prison constitue un programme ambitieux et un levier essentiel. Au 1 janvier 2024, dix neuf établissements ont déjà été livrés, et près de la moitié des établissements du programme immobilier seront opérationnels dès cette année.

omerta politique » : voilà ce qui restera du rapport sur le financement public de l’enseignement privé des députés Paul Vannier, du groupe

Notre Constitution pose un certain nombre de règles interprétées par le Conseil constitutionnel. Au nombre de celles ci figure le principe de la liberté d’enseignement, depuis 1977 comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cela signifie donc qu’aux côtés des établissements publics des établissements privés sous contrat

Bien sûr, j’aurais pu inviter ses détracteurs à sortir de la caricature et à trouver dans l’enseignement privé quelques clés de réussite, afin de redonner ses lettres de noblesse à l’enseignement public. Faites donc un rapport ! Je souhaiterais plutôt vous faire part d’une impression. Ceux qui, au nom de leur dogme, ont malmené l’école publique n’enragent ils pas désormais de constater, impuissants, la réussite de ceux qui ont gardé leurs distances avec certaines folies destructrices ? Est ce vraiment la faute de l’enseignement privé s’il n’a pas passé par dessus bord les concepts d’autorité, de mérite, de respect, de discipline, d’assiduité et d’excellence qui, pendant longtemps, ont fait les beaux jours de l’école publique ? Si l’école publique se portait mieux, l’école privée serait elle vraiment un problème pour eux ? Et l’éducation à la sexualité ? Devons nous, pour faire plaisir à quelques enragés, piétiner la liberté de choix des parents et détruire l’école qui fonctionne encore ? Mes chers collègues, allons nous vraiment les laisser faire ? La parole est à M. Jean Claude Tissot, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Plutôt que ce terrible retour en arrière, la France devrait encourager une révision de cette PAC, qui est à bout de souffle, qui ne protège ni les agriculteurs ni les consommateurs contre la forte volatilité des prix, et qui n’incite pas suffisamment à lancer l’indispensable transition agroécologique. il est essentiel de revoir le logiciel de la PAC, en commençant par le système des aides. Sortons des aides à l’hectare et au volume, pour passer à un système fondé sur l’actif agricole. Fixons un plafonnement pour assurer une meilleure répartition entre les agriculteurs, comme le fait déjà l’Espagne. Mettons en place un système d’aides contracycliques plafonnées permettant de dégager des moyens pour soutenir les filières en crise. Surtout, renforçons les mesures favorisant la transition agroécologique, avec des critères ambitieux et une valorisation des services environnementaux rendus par les paysans.

adapter son plan stratégique national pour permettre cette révision, contrairement à ce que nous a indiqué Mme la ministre déléguée Pannier Runacher à la fin du mois de février. Comptez vous, monsieur le ministre, profiter de cette occasion pour inclure des mesures qui permettront vraiment de remettre du revenu dans les fermes ? La parole

Comment réaliser ces 10 milliards d’euros supplémentaires sans autre texte financier ? D’abord, nous détenons plus de 7 milliards d’euros de réserve de précaution au sein des ministères, précisément

à l’heure où l’on apprend qu’en 2024 le déficit public de la France atteindra plus de 5 % du PIB au lieu des 4,4 % initialement prévus et qu’il faut donc faire des économies tous azimuts, le régime d’indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers interroge plus que jamais. En effet, selon le droit européen en vigueur, un Français domicilié en France qui perd son emploi dans un État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse est principalement indemnisé par l’Unédic.

Résultat : entre 2012 et 2020, les sommes déboursées par l’Unédic en raison de ce dispositif ont explosé. Elles sont passées de 540 millions à 920 millions d’euros par an,

parfaitement raison, et votre constat est totalement juste. Les règles d’indemnisation du chômage des frontaliers qui travaillent dans un pays de l’Union européenne ou en Suisse et qui résident en France

pour que l’État dans lequel la personne a travaillé prenne en charge l’indemnisation. Cela semble logique, mais, malheureusement, bon nombre d’États membres s’y opposent. Cette négociation, qui porte sur l’ensemble des volets de la sécurité sociale, dure depuis 2016.

que par respect pour les entreprises françaises et leurs salariés qui portent la charge de cette indemnisation du chômage des travailleurs transfrontaliers licenciés à l’étranger. Le financement de l’écart ne peut pas incomber à ces personnes et à ces entreprises. Les élections européennes constituent sans doute un moment opportun pour faire avancer ce sujet.

santé. Dans ce contexte de crise généralisée, le Gouvernement a annoncé, sans concertation ni dialogue, une hausse de 4,3 % des tarifs des hôpitaux publics, alors que le secteur privé lucratif devra, quant à lui, se contenter d’une hausse indigente de 0,3 Même si l’inflation est de 4 % pour tous, vous justifiez cet arbitrage inique en expliquant que le secteur privé a connu une forte dynamique ces dernières années. Or l’activité du secteur privé lucratif a servi à compenser la faiblesse de l’activité du secteur public. Contrairement aux idées reçues, les établissements de santé privés contribuent aussi à la prise en charge de patients précaires et sont parfois l’unique recours dans les déserts médicaux. Votre décision aggravera malheureusement une situation déjà critique, puisque les charges augmentent de façon exponentielle, tandis que les tarifs demeurent insuffisants pour assurer une gestion viable des établissements. En 2024, 50 % des établissements de santé privés seront en déficit, alors qu’ils représentent 35 % de l’activité hospitalière. Pour couronner le tout, le Premier ministre a annoncé, entre autres choses, l’expérimentation de la fin du parcours de soins et la revalorisation des séances de psychologues en accès direct, qui passeront de 30 euros à 50 euros. Parallèlement, dans le cadre des négociations conventionnelles avec l’assurance maladie,

à compter du 3 juin prochain. Les Français ne pourront pas continuer à être soignés sans les médecins libéraux et sans l’hôpital privé ! Allez vous donner des moyens au secteur privé lucratif, afin d’éviter à terme la fermeture d’hôpitaux privés ? Avez vous des propositions concrètes à faire pour soutenir les médecins libéraux ?

La parole est à M. Pierre Alain Roiron, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Vous n’avez cessé de vous en prendre à notre système social : réforme de l’assurance chômage, réforme des retraites, etc. Aujourd’hui encore, vous exprimez un mépris certain envers le cœur de notre service public, les fonctionnaires. Vous ne répondez pas à leur demande d’ouvrir de réelles négociations avec les partenaires sociaux, puisque vous ne proposez qu’une simple concertation, dont chacun connaît par avance le résultat : c’est la fameuse verticalité ! Vos propositions ?

c’est l’emploi à vie, qui permet d’éviter la concurrence salariale avec le privé et de limiter la corruption. Votre réforme ne répond pas aux préoccupations majeures

de vous répondre, permettez moi de saluer les agents publics de notre pays, ceux qui, dans nos écoles, nos commissariats, nos hôpitaux, nos collectivités territoriales, servent nos concitoyens et font vivre le service public, qui appartient à tous les Français.

pour la réplique. Selon le Premier ministre, « quand tu casses, tu répares ». Or, depuis 2017, vous avez beaucoup cassé : le système social, le système de soins, l’assurance maladie

de la jeunesse. Nul n’ignore le point commun entre Samuel Paty, Dominique Bernard et le proviseur du lycée Maurice Ravel : ils ont été lâchement assassinés par les terroristes islamistes ou bien contraints de démissionner. Combien se taisent et ont peur ? Nul n’ignore le sort de Mila.

vous avez indiqué qu’un enfant par classe était harcelé. Mes questions sont précises : combien de petits Français comme Samara ou Shemseddine sont ils menacés et harcelés pour une réputation aux allures de charia ? Ces situations sont elles précisément recensées dans votre bilan des signalements des atteintes à la laïcité et de harcèlement ? Si oui, quelles en sont les conséquences concrètes ? Enfin, que faites vous pour écarter vraiment les harceleurs, responsabiliser leurs parents et empêcher que l’islamisme poursuive la conquête de nos écoles ?

que la lutte contre le harcèlement sont des éléments sur lesquels nous sommes arc boutés. La laïcité, je l’ai dit à plusieurs reprises devant vous, est le terrain neutre permettant réellement aux enseignements fondés sur la science, et non pas sur ce que

pas à dire à quel point nous souhaitons vraiment que ces phénomènes de harcèlement cessent dans nos établissements.

Responsabilisation des parents, suspension des allocations familiales, port de l’uniforme, qui arrive tardivement et avec parcimonie, respect de la laïcité dans le sport, interdiction du port du voile pour les accompagnatrices scolaires, et tant d’autres mesures : pourquoi le Gouvernement s’y est il systématiquement opposé pendant des années ? Une fois encore, une fois de trop, nous voyons dans notre pays, non pas des « zones de non droit », mais des « zones d’un autre droit » dans lesquelles l’islamisme s’affiche en uniforme et menace nos enfants, nos enseignants et nos proviseurs, où les mœurs islamistes la police du vêtement se mêlent au harcèlement, où l’impunité l’emporte sur la fermeté, où la cruauté l’emporte sur l’autorité. La violence, le communautarisme et le radicalisme comblent le vide laissé par le refus de transmettre ce qui nous unit, le refus du commun, le refus de transmettre la culture et l’autorité.

Nous avons également proposé de revenir sur l’obligation de transfert des compétences eau et assainissement des communes aux communautés de communes, en autorisant un transfert direct et, donc, sans subdélégation desdites compétences des communes aux syndicats.

est reprise. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie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 J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

un déficit de 12 milliards d’euros, éventuellement envisageable dans douze ans, semblait gérable, sans que l’effort doive porter, brutalement et lourdement, sur les plus vulnérables. Depuis 2017, les retraités ont subi une baisse de leur pouvoir d’achat en raison de la hausse de la contribution sociale généralisée et de la sous indexation des pensions. Contrairement aux assertions alarmistes qui ont été celles du Gouvernement durant plusieurs mois, les comptes de notre système de retraite étaient équilibrés en 2023. La part de la richesse nationale consacrée aux retraites devrait ainsi rester stable dans les années à venir. Mais les Cassandre des retraites préfèrent évoquer le solde du système de retraites, les milliards d’euros ainsi affichés étant plus propices à affoler les Français… Il est pourtant démontré que l’expression en parts de PIB est bien plus efficace que celle en termes de solde, tant ce dernier peut être soumis à des variations aussi soudaines qu’imprévisibles.

Aujourd’hui, alors que la réforme est adoptée, on estime que notre système des retraites devrait revenir au quasi équilibre à l’horizon 2030. Mais, au delà de cette échéance, les effets de la réforme se dissiperont : à la réduction des dépenses issues d’une baisse du nombre de départs à la retraite devrait en effet succéder leur hausse du fait de l’augmentation de la durée des carrières

son PIB en 2023. Nous actons également le fait que, responsable de cette dérive du budget de l’État, le Gouvernement ne se décide pas à changer de cap ou de politique ni à modifier la manière dont il gère les finances du pays. Choisir de s’attaquer aux recettes de l’État en baissant les impôts des entreprises et des plus riches est un choix qui a pourtant fait l’éclatante démonstration de son inanité. Mais l’exécutif est très attaché à cette stratégie et ne souhaite pas y mettre un Il préfère inspecter les caisses des assurances sociales et tirer profit des petites machineries réglementaires et législatives qu’il a mises en place pour soustraire la gestion de ces dernières aux partenaires sociaux.

un milliard d’euros à l’association, contrainte de s’endetter pour satisfaire aux exigences du Gouvernement. Sans réelle politique de sauvegarde du système de protection des actifs, le Gouvernement ambitionne surtout de corriger le résultat budgétaire de ses choix politiques. Ce faisant, il met en péril le modèle de l’assurance chômage, pour renflouer d’autres caisses qu’il a très mal gérées. Ce n’est pas non plus pour sauver l’Agirc Arrco que le Gouvernement a essayé de prélever un milliard d’euros sur les fonds de cette caisse de retraite complémentaire cette dernière se porte bien, du fait de sa gestion rigoureuse par les partenaires sociaux. Et ce n’est pas non plus pour sauver le système des retraites que le Gouvernement a imposé sa réforme paramétrique de report de l’âge de départ. elle n’offre pas de solution de long terme pour la pérennité de notre modèle par répartition. En revanche, ce qui est sûr, c’est qu’elle a d’ores et déjà un coût social important. À moyen et long termes, le Gouvernement a créé des actifs particulièrement vulnérables, des seniors sans emploi ni retraite qui, âgés de 53 ans à 69 ans, n’ont déclaré au cours d’une année civile ni revenu d’activité ni pension de retraite, que ce soit en propre

au Conseil d’orientation des retraites, Michaël Zemmour estimait déjà à 300 000 le nombre de personnes supplémentaires qui seraient maintenues dans le sas de précarité entre emploi et retraite, en cas de report de l’âge légal

Loin de corriger le tir, l’exécutif a décidé d’agrémenter sa réforme des retraites de la suppression de l’allocation de solidarité spécifique, et d’acculer ces seniors à solliciter les départements, déjà débordés, pour bénéficier du RSA. Les travaux et auditions que nous avons menés depuis 2017 ont, en tout état de cause, mis en évidence le fait qu’aucun projet de réforme des retraites visant à faire travailler les gens plus longtemps ne peut être envisagé sans,, des mesures préalables en faveur de l’emploi des seniors et de prise en compte de la pénibilité. pénibilité. Madame la ministre déléguée, vous songez aujourd’hui à raboter les droits au chômage des seniors. Le Gouvernement prend le risque, ce faisant, de jeter des centaines de milliers de personnes dans la précarité, et met en péril l’équilibre budgétaire des collectivités territoriales chargées de l’insertion. Cette tentative pour masquer les conséquences de vos choix idéologiques et politiques ne trompe personne. De fait, les arguments que nous avons invoqués l’année dernière demeurent valables.

Le Gouvernement avait promis le retour à l’équilibre du système de retraite en 2030. Le COR l’a montré avec beaucoup de clarté : le système sera toujours déficitaire en 2030, à hauteur d’environ 5 milliards d’euros, et le restera d’ici à 2070, la réforme tendant même à accroître les dépenses de retraites à cet horizon.

Or, dans la foulée de la réforme, ceux ci ont non seulement rendu le cumul emploi retraite créateur de droits – comme c’est désormais le cas pour les régimes de base –, supprimé le bonus malus appliqué depuis 2019, qui avait perdu toute justification du fait du report de l’âge légal

Cette trajectoire n’est évidemment pas sans conséquence sur celle du système de retraite. Celui ci ne sera donc pas à l’équilibre en 2030, tant s’en faut, contrairement à ce qu’annonçait le Gouvernement pendant l’examen du texte.

affecte bel et bien la vie quotidienne des Français. À l’horizon de 2070, l’âge moyen de départ à la retraite sera relevé de six mois supplémentaires, pour s’établir à 64,6 ans.

au cours de l’année précédant la liquidation de leur pension, soit juste avant de partir à la retraite. Ils seront donc nécessairement maintenus dans cette situation du fait du relèvement de deux ans

pour chaque euro de dépenses économisé pour les retraites, 25 centimes supplémentaires seront dépensés au titre des autres prestations sociales.

Les femmes, en effet, bénéficient majoritairement des majorations de durée d’assurance accordées au titre de la naissance et de l’éducation des enfants. Ces trimestres leur permettent, en règle générale, d’atteindre plus tôt que les hommes la durée d’assurance requise pour le taux plein, ce qui contribue à expliquer que l’âge moyen de départ à la retraite des femmes soit légèrement inférieur à celui des hommes. Or, du fait du report de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite, les majorations de durée d’assurance seront en quelque sorte « écrasées » par des trimestres cotisés, et les deux années de travail supplémentaires L’exemple de la génération de 1972 est emblématique de cette injustice frappante : les hommes de cette génération partiront en moyenne cinq mois plus tard qu’avant la réforme,

La revalorisation de 100 euros des minima de pension, mise en avant avec insistance par le Gouvernement, devait garantir aux travailleurs une retraite minimale de 1 200 euros par mois. La réalité est malheureusement bien différente. D’après la Caisse nationale d’assurance vieillesse, le montant accordé aux nouveaux retraités au titre du minimum contributif n’a augmenté que de 30 euros en moyenne en 2024. Les personnes parties à la retraite avant l’entrée en vigueur de la réforme devaient, pour leur part, bénéficier d’une majoration exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 100 euros. Or seuls 20 000

réforme, qui a fait l’objet de quatre mois de concertation et de 175 heures de débats parlementaires, est allée au bout de son cheminement démocratique. Aujourd’hui encore, le Gouvernement défendra cette réforme indispensable pour assurer l’avenir de notre système par répartition, qui est pleinement entrée en vigueur depuis le 1 septembre dernier.

inadmissible ! Le Gouvernement s’y opposera sans surprise. Vous voulez abroger purement et simplement la réforme des retraites de 2023, alors qu’elle est déjà entrée en vigueur. Concrètement, qu’est ce que cela signifie ? d’aggraver de près de 14 milliards d’euros le déficit de notre système de retraite en 2030 et de supprimer la revalorisation des petites pensions : pour 185 000 nouveaux retraités chaque année, cela signifie 30 euros de plus chaque mois. Mais, pire encore, pour 550 000 petites pensions ayant déjà été liquidées, c’est une revalorisation moyenne de 50 euros par mois qui s’applique depuis septembre dernier.

Sur ce point, nous n’évitons pas le débat et nous rappelons ce qui a motivé notre choix de faire travailler progressivement plus longtemps les Français qui le peuvent.

Cette assemblée a régulièrement défendu une augmentation encore plus rapide de l’âge légal de départ. Travailler plus longtemps, c’est enfin le moyen le plus juste de financer les progrès et les avancées de la réforme. Ce qui est au cœur de notre désaccord et, donc, au cœur de votre proposition est au fond assez simple : au premier alinéa de l’article unique, vous proposez de revenir sur la réforme des retraites.

Quant à la simplification des contraintes qui pèsent sur les entreprises, nous y travaillons : le ministre de l’économie présentera prochainement un projet de loi de simplification de la vie des entreprises, et la ministre du travail présentera également un projet d’acte II de la réforme du marché du travail, qui simplifiera la vie des employeurs.

Monsieur le président, madame la ministre

sans précédent du débat parlementaire, avec la complicité de la droite des deux assemblées. C’est un passage en force antidémocratique sous couvert de sauvegarde du régime des retraites

que l’ensemble des régimes présenteront un besoin de financement de 0,2 à 0,3 point de PIB à cette échéance, soit 5 à 8 milliards d’euros. Cette réforme est déjà frappée d’inefficacité, car elle reposait sur des hypothèses macroéconomiques

et des effectifs des fonctionnaires, à la sous compensation de certaines exonérations de cotisations sociales, à la multiplication des primes désocialisées dont l’effet substitutif est prouvé, à la déflation salariale, ainsi qu’à certaines mesures de la réforme des retraites pense aux modifications apportées au cumul emploi retraite, qui augmentent le coût d’un dispositif favorisant l’allongement du temps de travail. Nous avons en revanche soutenu

même si la revalorisation des pensions n’est que de 30 euros en moyenne. Rappelons le, ce n’est que l’application d’une promesse liée à la précédente

Il y a un peu plus d’un an, le 11 mars 2023, le Sénat achevait l’examen de la réforme des retraites. Le 14 avril de la même année, le Conseil constitutionnel validait officiellement le recul social le plus grave de la décennie.

Lorsque nous avons appris le dépôt par le groupe socialiste, le 26 février 2024, d’un texte similaire, nous nous sommes rassemblés dans un pôle progressiste contre le Gouvernement et la majorité sénatoriale. C’est avec un certain plaisir que nous avons entendu la majorité sénatoriale reconnaître, la semaine dernière, que cette réforme, dont elle a toujours revendiqué la paternité, s’inscrivait dans une logique purement budgétaire. Le président Bruno Retailleau s’était personnellement impliqué pour faire voter l’allongement de la durée de cotisation à quarante trois annuités et le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, au nom de la préservation de notre système de retraite par répartition.

D’un côté, les salariés doivent accepter des sacrifices sur leurs droits collectifs au nom du maintien de l’équilibre du système de retraites. De l’autre, mes chers collègues de droite, vous agissez pour développer la capitalisation individuelle et les fonds de pension américains, si chers à vos cœurs. aux accents de déjà vu offre l’occasion au Gouvernement et à la majorité sénatoriale de justifier une réforme injuste, inefficace et inégalitaire. Vous allez nous rejouer le débat sur les retraites sur l’air de l’austérité et du dérapage des dépenses publiques. Je rappelle que le déficit des retraites à l’origine de votre réforme scélérate

Le démantèlement des « conquis sociaux » se fait au détriment de la prise en compte de la pénibilité des métiers. La suppression des régimes spéciaux, qui permettaient une meilleure prise en considération de la réalité des conditions de travail, est une perte immense immense pour les cheminots, les électriciens, les gaziers et les salariés des autres régimes fermés. En faisant le choix d’accélérer le calendrier de la réforme Touraine, le Gouvernement s’est attaqué aux plus précaires. L’augmentation de la durée de cotisation frappe en premier lieu les femmes ayant des carrières hachées, les salariés aux métiers pénibles et les personnes ayant fait des études longues. En maintenant la décote sur les pensions incomplètes, vous avez aggravé la précarité tout en préservant les intérêts des plus riches et des puissants. La droite sénatoriale et le Gouvernement ont systématiquement

nous défendons un projet solidaire où l’humain prime la finance et les intérêts des multinationales. Vous avez fait adopter un projet brutal, en recourant au 49.3 après des mois de mobilisation sociale.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

un goût amer à tous ceux qui en avaient compris les enjeux : financer les prochaines retraites dans un contexte de vieillissement démographique, mais surtout de désenchantement du monde professionnel. Le groupe du RDSE a toujours défendu une réforme du système des retraites, qui consisterait à remplacer les annuités par des points au sein d’un régime universel. Les rapports du COR ont souvent démontré qu’une telle mesure était techniquement possible et permettrait notamment d’intégrer des dispositifs de solidarité. C’était d’ailleurs la réforme proposée par le Président de la République en 2019, avant qu’il ne l’abandonne en raison de la crise de la covid 19 et des contestations sociales. Mais pas de débat non plus à ce sujet Le Gouvernement n’a donc prévu qu’une anticipation de la loi Touraine et le report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans. L’éléphant a accouché d’une souris ! Ce seul changement n’aurait pas dû enflammer la sphère politique qui, avec raison et conscience, depuis des décennies, du président Sarkozy au président Hollande, a toujours pris ses responsabilités pour réformer le régime des retraites et son équilibre. Revenir aujourd’hui avec cette proposition de loi pour modifier ce seul indicateur d’âge, c’est légiférer pour légiférer, moins d’un an après

avec une augmentation notable des absences chez les plus jeunes. Deux indicateurs sont particulièrement inquiétants : les maladies professionnelles, principalement les troubles musculo squelettiques, ainsi que les pathologies psychologiques sont à l’origine des arrêts de travail dont la durée est la plus longue. L’enjeu crucial qui devrait nous animer est celui du bien être au travail. Nous devons penser au delà des querelles politiques pour avancer. Prenons les problèmes à bras le corps. Si le contexte nous a obligés, dès 2013, à envisager une durée de travail de 43 ans, unissons nous pour le bien être des travailleurs

tout le monde nous l’envie : notre système de retraite par répartition, fondé sur la solidarité intergénérationnelle, est un système unique, fierté de notre nation. Le principe est simple : les cotisations des actifs servent à payer les pensions des retraités. C’est un système d’équilibre qui, si une génération n’y trouve pas son compte, peut s’effondrer. Cet équilibre a pour socle l’évolution démographique. En 1980, il y avait 2,68 actifs pour un retraité, contre 1,67 en 2020. Et en 2050, il n’y aura plus qu’environ 1,3 actif pour un retraité. Le socle se dégradant, nous ne pouvions rester les bras ballants. Trois leviers étaient à notre disposition pour maintenir le système à l’équilibre : augmenter les cotisations des actifs, diminuer les pensions des retraités ou augmenter le nombre d’années travaillées par les actifs. On pourrait en imaginer un quatrième, j’y reviendrai. Le Gouvernement, suivi par sa majorité, ainsi que par celle du Sénat, a pris la décision d’utiliser l’allongement de la durée du travail comme levier qui, si je ne m’abuse, s’inscrit dans la même veine que la réforme proposée par Mme la ministre Touraine.

Sauf erreur de ma part, les socialistes, alors majoritaires, et leurs alliés – à l’exception des communistes – l’ont soutenue sans réticence. De fait, il s’agissait d’un vote relativement indolore, puisque ses effets ne se feraient sentir qu’au delà de leur mandat Pour notre part, nous avons pleinement assumé notre réforme et son application immédiate, tout en l’améliorant pour protéger les plus vulnérables. C’est une blague ? Ça s’est vu dans la rue ! Nous nous retrouvons aujourd’hui, à la demande de ceux qui ont soutenu la réforme Touraine, pour abroger un texte qu’ils auraient pleinement approuvé en 2014 : Kafka, sors de cet hémicycle

n’est cependant pas la seule et unique conséquence, et je m’étonne que mes collègues socialistes, auteurs de cette proposition de loi, et si prompts à revendiquer les valeurs sociales, n’en aient pas parlé. Vous qui vous réclamez des valeurs fondamentales que sont l’égalité et la solidarité, comment récupérez vous les 6,8 milliards d’euros de mesures qui accompagnent la réforme que vous nous proposez d’abroger ici et maintenant ?

À l’heure où la défiance envers les responsables politiques se fait de plus en plus vive, nous devons réaffirmer notre devoir : dire la vérité aux Françaises et aux Français. Oui, certaines des mesures

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour débattre de la proposition de loi du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visant à abroger la réforme des retraites adoptée il y a un an. Permettez moi de rappeler les circonstances dans lesquelles cette réforme a été adoptée. Malgré l’opposition des syndicats et des manifestations d’une ampleur sans précédent, le Gouvernement s’est obstiné à faire passer cette réforme à marche forcée. En ayant recours à un projet de loi de financement rectificative

exprimée, voire pas du tout. Le Gouvernement a également fait usage du vote bloqué prévu à l’article 44.3 de la Constitution pour contraindre les sénateurs à se prononcer sur le texte par blocs d’amendements, sélectionnés par lui même. Ce faisant, il a ignoré l’avis des partenaires sociaux, bafoué le rôle du Parlement, saboté le débat parlementaire et précipité une réforme profondément injuste. Les conséquences de cette réforme ne sont pas digérées. La justification avancée par le Gouvernement pour le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans reposait sur la réduction du déficit, avec la promesse d’un système équilibré d’ici 2030. On en sera loin ! Décidément, les prévisions du grand argentier de l’État, M. Le Maire, ne font pas recette ! Loin d’équilibrer notre système de retraite, cette réforme a des conséquences économiques et sociales dégradées sur des catégories déjà fragilisées. Le relèvement de l’âge d’ouverture des droits entraîne une augmentation des coûts pour notre protection sociale. La direction générale du Trésor prévoit une hausse d’environ 3,2 milliards d’euros des dépenses sociales

ce n’est pas de la communication ! Avec de telles prévisions, on comprend mieux l’empressement du Gouvernement à vouloir réformer l’assurance chômage et supprimer l’ASS ! Cette réforme injuste pénalise particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui occupent souvent les métiers les plus pénibles.

et ne perçoivent donc pas leur retraite. Cette réforme fait abstraction de la question de la pénibilité, ce qui est d’autant plus préoccupant que quatre des dix critères de pénibilité ont été supprimés par les ordonnances Travail de Muriel Pénicaud. Les travailleurs seniors sont particulièrement pénalisés, la grande majorité des personnes au chômage à l’âge de 60 ans n’ayant pas l’occasion de retrouver un emploi. Alors que les mesures timides pour améliorer l’emploi des seniors ont été invalidées par le Conseil constitutionnel, le Gouvernement a choisi de reporter ce sujet à des négociations ultérieures, changeant ainsi l’ordre des priorités : d’abord une réforme drastique, puis des discussions sur la manière dont les personnes concernées pourront travailler deux années de plus. Plutôt que d’encourager les entreprises à recruter ou à maintenir les seniors en poste, le Gouvernement multiplie les annonces de réduction des droits, notamment en matière de chômage, comme si le fait de rester sans emploi relevait d’un choix volontaire. Les femmes sont également les grandes perdantes de cette réforme. En règle générale, elles atteignent plus souvent que les hommes la durée de cotisation requise à l’âge de 62 ans, en raison des majorations de durée d’assurance accordées pour la maternité et l’éducation des enfants. Le report de l’âge légal à 64 ans les oblige à prolonger leur activité de deux années supplémentaires sans bénéficier d’avantages significatifs, tandis que les hommes sont souvent déjà contraints de travailler au delà de 62 ans pour obtenir une retraite à taux plein et sont donc moins affectés par cette disposition. En ce qui concerne l’une des principales mesures d’accompagnement de la réforme, consistant à augmenter de 100 euros le minimum contributif des régimes alignés et la pension majorée de référence (PMR) du régime des non salariés agricoles, elle ne profite en réalité qu’à une infime partie des assurés. En effet, seuls ceux qui ont cotisé tout au long de leur carrière au niveau du salaire minimum sont censés bénéficier de cette augmentation de 100 euros. Malheureusement, les bénéficiaires sont peu nombreux. Quelle déception pour ceux qui avaient cru en cette revalorisation ! Des solutions existent pour assurer la pérennité de notre système de retraite. La question des recettes ne doit pas être un tabou. Selon les estimations de la direction de la sécurité sociale, une augmentation d’un point du taux de la cotisation patronale d’assurance pourrait générer des recettes estimées à 6,8 milliards d’euros si elle ne touchait que l’assiette plafonnée. Par ailleurs, la suppression partielle des allégements généraux de cotisations sociales, qui représentent une perte de près de 60 milliards d’euros de recettes pour la sécurité sociale en 2022,

Enfin, la création d’une taxe sur les superprofits – une proposition récemment soutenue par la présidente de l’Assemblée nationale – est une piste qui pourrait également être explorée. Mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain continue de s’opposer à cette réforme brutale aux effets délétères. Je tiens donc à saluer le travail accompli par mon groupe,

Nos collègues socialistes proposent en effet d’abroger purement et simplement la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, qui porte la dernière réforme des retraites. Au delà de l’affichage politique et dogmatique, prenons quelques minutes pour rappeler en quoi revenir sur cette réforme serait une folie. Être parlementaire, mes chers collègues, c’est d’abord faire preuve de responsabilité.

et celles de leurs enfants seront financées. Notre responsabilité n’est pas d’ignorer les difficultés ou de laisser à nos successeurs le soin de les régler. Au contraire, elle nous invite à regarder la situation en face et à lui apporter des réponses durables et justes. Chacun sait ici que, pour financer les retraites, il y a trois voies possibles. La première est de baisser les pensions des retraités. Nous nous y refusons, car, du fait de leur indexation sur l’inflation, le niveau de vie moyen des retraités devrait passer de 101 % du niveau de vie des actifs en 2019 à 85 %, voire 75 % en 2070. La deuxième est d’augmenter massivement les cotisations ou la fiscalité. Nous nous y refusons également, car les prélèvements obligatoires représentent déjà 48 % de notre PIB, soit le record de la zone euro. Relever le taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse, comme le suggère Mme la rapporteure, accroîtrait le coût du travail et fragiliserait encore davantage la compétitivité des entreprises françaises.

C’est la voie la plus raisonnable, celle que tous les autres pays ont choisie et que nous avons retenue, car nous vivons plus longtemps : depuis 1950, notre espérance de vie Rappelons qu’avant la réforme de 2023 l’âge légal de départ à la retraite de la France était l’un des moins élevés des pays de l’OCDE. Après le relèvement à 64 ans, il reste en dessous de celui de nombreux autres pays il est de 65 ans en Belgique, à Chypre ou en Espagne, et s’élève même à 67 ans en Allemagne, en Italie ou au Danemark. Je pose donc la question à nos collègues socialistes : pourquoi vous opposez vous aujourd’hui au report de l’âge légal à 64 ans après l’avoir voté en 2014 ? ? Faut il vous le rappeler ? Même sans la réforme de 2023, l’âge moyen de départ à la retraite devait de toute façon atteindre les 64 ans dans le courant des années 2030 du fait des réformes allongeant la durée de cotisation,…

Au delà de la question démographique, le contexte budgétaire paraît particulièrement mal choisi pour renoncer aux recettes générées par la réforme de 2023. de la sécurité sociale pour 2024 souligne que, malgré cette réforme, une dégradation de la trajectoire financière de la branche vieillesse s’annonce. D’ici à 2027, le déficit de cette branche pourrait s’établir à 11,2 milliards d’euros en raison, notamment, du vieillissement démographique, du ralentissement de la croissance de la masse salariale du secteur privé et des difficultés financières du régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. sans la réforme des retraites de 2023, le déficit de la branche vieillesse serait de 17,5 milliards d’euros en 2027. Réformer les retraites, c’est donc empêcher une nouvelle dégradation des comptes publics. C’est aussi se donner la possibilité d’augmenter le taux d’emploi des seniors pour créer des recettes autres que des cotisations vieillesse pour un montant qui pourrait atteindre, selon la direction générale du Trésor, 15 milliards d’euros par an. Enfin et surtout, en voulant abroger le texte de 2023, vous abrogez la réforme dans son intégralité, y compris tous les apports que le Sénat avait obtenus, parfois de haute lutte, et sur lesquels il paraît aujourd’hui inconcevable de revenir. En abrogeant cette réforme, vous abrogez la création de l’assurance vieillesse des aidants, la revalorisation des minima sociaux, la création de la pension d’orphelin et de la surcote de 5 % pour les mères qui ont validé leur durée d’assurance. Vous abrogez aussi les nouveaux droits en matière de carrières longues qui profitent déjà aux Français : à la fin de l’année 2023, 30 % des nouveaux retraités concernés par la réforme sont partis avant l’âge légal grâce à ce dispositif, contre 20 % fin 2022, selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Je pourrais aussi évoquer les apports visant à prendre en compte l’engagement des citoyens, comme l’octroi de trimestres pour les sapeurs pompiers volontaires ou encore la possibilité pour les élus locaux de cotiser intégralement sur leurs indemnités. Je citerai enfin le renforcement de la lutte contre la fraude, avec notamment des contrôles biométriques de l’existence des pensionnés résidant à l’étranger mis en place à compter de la fin de l’année 2023. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, la réforme telle que nous l’avons votée est la seule voie possible pour sauver notre système de retraite. Bien sûr, elle n’est pas parfaite. Nous aurions voulu aller plus loin, notamment sur l’emploi des seniors. Mais n’oublions pas tout le travail réalisé par le Sénat pour améliorer la version initiale du Gouvernement. Plutôt que de vouloir abroger cette réforme et imaginer des scénarios alternatifs non réalistes, concentrons nos efforts sur une nouvelle loi Travail et sur l’accompagnement des salariés, en améliorant la prévention en matière de santé et la sécurité, afin que ceux ci soient toujours en bonne santé au moment de prendre leur retraite. Pour conclure, cette proposition de loi est symptomatique du décalage entre les discours de la gauche française et la réalité du monde dans lequel nous vivons. À chaque fois qu’elle s’est retrouvée au pouvoir, elle a, par ses réformes, laissé croire aux Français qu’ils pourraient travailler moins longtemps, à rebours de tous les autres pays ayant une économie comparable. Cela a commencé avec l’abaissement de l’âge de départ à la retraite de 65 à 60 ans voulu par François Mitterrand. Cela a continué sous le gouvernement de Lionel Jospin avec les 35 heures de Mme Aubry, une idée tellement lumineuse qu’aucun autre pays au monde n’en a voulu ! Le groupe Les Républicains ne laissera pas dénaturer la réforme de 2023, car ce serait mettre en péril le retour à l’équilibre de notre Notre principal objectif est bien de sauver notre régime par répartition et de garantir ainsi à nos concitoyens que le pacte social conclu après guerre restera toujours bien vivant.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, deux ans après avoir fait réélire Emmanuel Macron, les socialistes semblent vouloir se racheter auprès de nos compatriotes en proposant un texte certes salutaire, mais dont ils savent qu’il n’aura aucune chance de l’emporter, ici comme à l’Assemblée nationale. La gauche semble tout d’un coup prise d’un certain remords. Pour autant, ce petit coup parlementaire ne saurait tromper personne et les classes populaires ont compris depuis longtemps ce Quant à la droite, nous regrettons qu’elle se soit ralliée aux discours trompeurs des libéraux, notamment au fameux argument « tarte à la crème » selon lequel, puisque l’on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps, en omettant toujours de dire que l’on ne vit pas plus longtemps en bonne santé, d’autant que la pénibilité a été, comme les carrières longues, la grande absente des débats l’année dernière ; le fils d’ouvrier, petit fils et arrière petit fils de mineur que je suis ne peut que le déplorer La majorité sénatoriale appelle à la responsabilité, nous dit que la situation financière dramatique impose un effort de nos compatriotes, mais, vous vous en doutez, si nous partageons ce constat, nos solutions d’économies sont grandement différentes et le recul de l’âge de départ à la retraite n’en fait pas partie. Pour finir ce tour d’horizon des responsabilités respectives, nous ne pouvons oublier le Gouvernement, naturellement. Alors qu’il a été porté au pouvoir sur une promesse de sérieux et de bonne gestion financière, la réalité a malheureusement éclaté au grand jour. Notre système de retraites n’a pas été sauvé par cette réforme. Pis, le Conseil d’orientation des retraites prévoit d’ores et déjà un déficit du système de retraites pour 2027, annonçant une réforme de plus grande ampleur et des économies supplémentaires, soit un nouveau tour de souffrances pour nos compatriotes. Pour autant, reconnaissons à Emmanuel Macron qu’il n’a trahi personne avec cette réforme ; il l’avait annoncée dans son programme en 2022 et tous ceux qui l’ont soutenu ici l’ont fait en connaissance de cause. Des économies à faire, il y en a. En premier lieu, nous pourrions nous attaquer au coût, sans cesse plus lourd, de l’immigration et de l’insécurité ou à la contribution nette, beaucoup trop nette, au budget de l’Union européenne. Alors, de grâce, cessons de vouloir saigner toujours plus nos compatriotes ! Si nous ne défendons pas un fumeux « droit à la paresse », nous défendons un droit au repos après des décennies de travail et de contribution aux finances de la France. La retraite, socle de notre pacte social, doit être profondément réformée. Il faut davantage soulager ceux de nos compatriotes qui effectuent les carrières les plus pénibles. La proposition présidentielle de Marine Le Pen reste donc toujours valable. Toutes les personnes qui auront commencé à travailler avant 20 ans pourront partir à la retraite à partir de 60 ans si elles ont 40 annuités de cotisation. Ceux qui ont commencé progressivement, après 20 ans, iraient jusqu’à l’âge de 62 ans. Voilà une réforme juste, nécessaire et utile pour nos compatriotes ! C’est la raison pour laquelle nous voterons cette proposition de loi, justement parce que nous ne sommes pas sectaires : dès lors

formation accentuée et, enfin, l’augmentation des petites retraites. En France, 57 % des travailleurs âgés de 55 à 64 ans sont en emploi, contre 72 % en Allemagne. L’objectif est donc d’augmenter le nombre de cotisants de 10 %, afin d’équilibrer le régime des retraites en 2030. Mes chers collègues, développer l’emploi des seniors sans précarité pour eux, afin d’équilibrer le régime et de maintenir les retraites par répartition, devrait être un objectif social commun pour nos enfants et l’avenir de la France. Cet objectif est visé par notre pays.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, en application de l’article 40 de la Constitution, selon lequel « [l]es propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique », le Gouvernement considère que la proposition de loi d’abrogation de la réforme des retraites portant l’âge légal de départ à 64 ans, présentée par Mme Monique Lubin et plusieurs de ses collègues, n’est pas recevable et ne peut donc pas être soumise à discussion. Refus

en application de l’article 45 du règlement du Sénat, l’irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée par la commission des finances. Quel est l’avis de la commission des finances

Monsieur le président, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 38 de notre règlement,

Je pense que l’examen de ce texte est nécessaire, ne serait ce que pour tirer un premier bilan de la réforme des retraites. Effectivement, celle ci fait débat, ce qui est parfaitement légitime. L’amélioration de la retraite des femmes, nos collègues ont dit tout à l’heure ce qu’il en était ; l’amélioration du taux d’emploi des seniors, qui devait accompagner cette réforme des retraites, nous voyons aujourd’hui ce qu’il faut en

par les groupes minoritaires. Nous défendons ici, au delà de la « niche » de nos collègues socialistes, le droit d’initiative parlementaire, prévu à l’article 45 45 de la Constitution. Jusqu’à présent, au Sénat, les propositions de loi étaient protégées de l’épée de Damoclès de l’article 40.

s’autodissoudre. Nous connaissons l’état des rapports de force au Sénat, donc nous connaissons déjà l’issue d’un vote sur l’abrogation de la réforme des retraites. Dès lors, pourquoi voulez vous empêcher le débat et le vote du Sénat ?

aux 70 % de Français qui étaient opposés à cette réforme, à ceux qui étaient dans la rue, et qui, depuis un an, digèrent très difficilement ce qui s’est passé l’année dernière. Madame la ministre, vous avez brandi l’article 40. Enfin, ce gouvernement dialogue avec le Parlement et prend une initiative ! Depuis trois mois

il y a vraiment besoin, dans ce pays, de faire de la politique pour parler aux couches populaires

pas de panique : ayez confiance en vos collègues de la commission des finances. Celle ci va se réunir et tout va bien se passer.

Allons au bout du débat, celui ci sera apaisé, respectueux et tout le monde aura sa légitimité pour donner son avis. La

La séance est reprise. Mes chers collègues, je vous rappelle que, en application de l’article 45 du règlement du Sénat, l’irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée par la commission des finances. Quel est l’avis de la commission des finances ? Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des finances s’est réunie et a estimé que la proposition de loi était irrecevable au titre de l’article 40

la parole est à M. Patrick Kanner, auteur de la proposition de loi.

par le poids des crises à répétition, le socle même de notre République, le lien social, est aujourd’hui mis à l’épreuve. C’est dans ce contexte tumultueux que je m’adresse à vous comme législateur, mais aussi comme défenseur d’une génération en quête de sens, de direction et surtout d’actions concrètes. La jeunesse française, animée par un désir d’engagement, pleine d’idéaux et de causes à défendre, se heurte pourtant à un mur de frustrations en raison d’un manque de possibilités et de moyens, ainsi que d’une confiance en l’avenir érodée. Devant cette réalité, des questions demeurent. Comment allons nous répondre à l’appel de nos jeunes ? Sommes nous prêts à transformer leur aspiration en une force motrice pour notre République ? La réponse – j’en suis convaincu, mes chers collègues – réside en partie dans le renforcement du service civique.

la solidarité, la conscience collective, la diversité des expériences sociales ainsi que le développement d’aptitudes favorisant l’insertion professionnelle. Ces aspects, qui sont au cœur de son action, en font un pilier essentiel dans le tissu socio éducatif de notre pays. Au fil des ans, le service civique s’est révélé être un vecteur d’orientation pour les jeunes, leur offrant souvent les clés pour affiner leur projet de vie professionnelle. négligé depuis 2017 au profit d’un dispositif inspiré de la culture militaire, par ailleurs tout à fait respectable. Pour notre part, nous préférons vous proposer un dispositif citoyen, ancré dans l’éducation populaire. Laissons derrière nous la nostalgie pour redynamiser ce dispositif éprouvé et transpartisan. Il est essentiel de se souvenir que l’engagement doit résulter d’un choix personnel. ci ne doit pas être imposé par le Gouvernement ; il doit émerger spontanément, comme le fruit d’une décision individuelle. Dans le contexte actuel de tensions, exacerbées par une jeunesse désorientée parfois jusqu’à l’extrême, comme l’ont cruellement illustré les émeutes de juillet dernier,

Animé par cette conviction, j’ai conçu une proposition de loi ambitieuse, articulée autour de cinq axes stratégiques, visant à augmenter considérablement l’attractivité et l’impact de ce dispositif. Mon objectif, qui est aussi celui du groupe socialiste, est clair : transformer positivement l’accès, la visibilité et la valeur de cet engagement dans la vie de nos jeunes. Premièrement, en élargissant l’accès au service civique jusqu’à 30 ans, nous ouvrons grand les portes de l’engagement. Cependant, étant conscient des questionnements autour d’une telle démarche, je salue la proposition pragmatique de Mme la rapporteure Sylvie Robert, qui limite cet élargissement à 27 ans, comme un premier pas mesuré et prometteur. Mais la recherche permanente du compromis m’amènera à vous proposer que l’élargissement puisse être expérimenté pour une période de trois ans. Deuxièmement, diversifier les structures d’accueil en y incluant les institutions de la République, c’est offrir une pluralité d’engagements possibles, garantissant ainsi à chaque jeune de trouver une mission qui lui ressemble.

Intégrer la possibilité d’effectuer un service civique au cœur du parcours académique, grâce à une année de césure assortie de la promesse d’un retour garanti en formation, marque un pas significatif vers une incorporation harmonieuse de ce dispositif dans nos trajectoires éducatives. Quatrièmement, revaloriser l’indemnité du service civique, qui reste largement en dessous du seuil de pauvreté, constitue une mesure de bon sens et un signal fort de notre engagement envers la jeunesse. Rappelons nous que les 18 25 ans sont les plus exposés à la précarité. L’indemnité actuelle de 620 euros, avec 505 euros 115 euros à la charge de l’organisme d’accueil, constitue un frein majeur pour de nombreux jeunes issus de milieux défavorisés. Une revalorisation de cette indemnité est impérative, afin de permettre à toutes les personnes désireuses de s’engager de le faire sans craindre pour leur subsistance financière. Cette problématique étant délaissée par l’exécutif pour des raisons comptables – je n’y reviens pas, cela a déjà été évoqué il nous incombe, à nous parlementaires, de prendre nos responsabilités pour permettre à toute cette génération de s’engager dignement. Cinquièmement, valoriser cet engagement dans les parcours académiques et professionnels, comme Parcoursup ou encore les concours de la fonction publique, c’est donner de la valeur à l’engagement et envoyer un message clair : la République reconnaît, valorise et récompense le service qu’ont rendu de jeunes citoyens. Mes chers collègues, ce que ce que vous propose le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, ce n’est pas seulement une réforme, c’est un appel à l’action, un appel à donner à notre jeunesse les moyens de s’engager malgré cette initiative législative, de nombreux défis restent à relever. Des interrogations subsistent, y compris au sein de mon camp politique au sens large. Originellement imaginé comme un engagement accessible à tous, sans exigence de compétences spécifiques, le service civique se trouve désormais à la croisée des chemins. Les pratiques condamnables telles que l’emploi déguisé ou la sélection sur compétences menacent son intégrité et son objectif d’inclusion, favorisant ainsi une certaine forme d’élitisme au détriment de la diversité sociale.

De plus, un renforcement du soutien aux structures d’accueil et aux tuteurs, une formation adéquate, un accompagnement continu et une augmentation des ressources financières et humaines à leur disposition est nécessaire pour assurer un encadrement de qualité pour les volontaires, dans le respect des principes fondateurs du service civique.

qu’à percevoir le revenu de solidarité active (RSA) –, que le Gouvernement et la majorité sénatoriale voient manifestement d’un mauvais œil, des mesures complémentaires telles que la prise en charge des frais de transport ou l’attribution d’un logement étudiant pourraient être envisagées pour éliminer les barrières matérielles à l’engagement. Seule une détermination continue à améliorer et à élargir le service civique fera de ce dispositif un véritable instrument d’émancipation et d’intégration sociale pour tous les jeunes, quelles que soient leur origine ou leur situation économique. Le service civique est une politique publique vertueuse. Mes chers collègues, l’heure est venue d’agir avec courage et conviction. Faisons du service civique la pierre angulaire d’une République bienveillante et empathique, une République qui écoute, qui inspire et qui valorise de jeunes citoyens. Unissons nous pour transformer le service civique en un pilier de notre cohésion nationale, un catalyseur pour une génération prête à affronter positivement les défis si lourds de notre époque. C’est bien ensemble que nous bâtirons une France plus forte, plus unie et infiniment plus inclusive, en faisant confiance aux jeunes générations ! La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une « école de l’engagement citoyen à davantage valoriser » : telle est la description du service civique faite de manière consensuelle par la mission d’information visant à renforcer la culture citoyenne de nos collègues Henri Cabanel et Stéphane Piednoir. Depuis la création du service civique, le nombre de volontaires n’a cessé de progresser. Après une phase d’expansion entre 2010 et 2017, le nombre annuel de missions se stabilise désormais autour de 80 000 par an. Au delà de ces chiffres, le service civique a su trouver sa place en tant que politique publique en faveur à la fois de la jeunesse et de l’engagement. Il a su convaincre également au sein de la classe politique, je tiens à le signaler : le service civique, issu d’une proposition de loi sénatoriale, traverse les courants politiques. Il a été mis en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est monté en puissance sous celle de François Hollande et a été officiellement intégré au sein du dispositif « 1 jeune, 1 solution » par Emmanuel Macron. Chaque année, ce sont des jeunes aux parcours très différents en termes d’âge, de diplôme, de situation ou d’origine qui deviennent volontaires. Cette variété des profils témoigne de la capacité du dispositif à remplir sa mission d’accueil de la jeunesse dans sa diversité pour constituer un moment de mixité sociale et d’engagement au service des autres. La proposition de loi de M. Kanner et du groupe socialiste vise à renforcer le service civique. Je salue cette initiative, qui va permettre au Sénat de souligner, de manière transpartisane – j’en suis convaincue –, l’utilité du dispositif, dans un contexte budgétaire qui s’annonce en revanche compliqué compliqué pour l’Agence du service civique : l’annulation de 100 millions d’euros de crédits est en effet évoquée… Au delà de ces perspectives budgétaires inquiétantes, de multiples obstacles subsistent, auxquels cette proposition de loi souhaite répondre. Tout d’abord, cette forme d’engagement est encore trop souvent méconnue des jeunes. Au cours de ses travaux, la commission de la culture a sécurisé le mécanisme de césure pour les jeunes en prévoyant dans la loi le droit de réintégrer la formation dans laquelle ils étaient inscrits avant leur mission. En effet, le service civique intervient le plus souvent lors des études supérieures, l’âge moyen des volontaires étant de 21 ans. En revanche, elle a supprimé l’obligation d’intégrer cet engagement parmi les critères devant être pris en compte dans l’examen des candidatures dans les filières sélectives. sélectives. Cela, vous l’imaginez, risquait de créer une rupture d’égalité. Autre obstacle identifié, l’indemnité, dont le montant constitue parfois un frein pour le jeune en situation précaire. Un premier effort a été fait voilà quelques mois pour porter l’indemnité à 620 euros, soit un montant supérieur au RSA. En accord avec l’auteur du texte, qui souhaite une augmentation supplémentaire de celle ci, j’ai proposé à la commission de l’aligner sur la rémunération touchée par un jeune de 18 ans en première année d’alternance. Nous aurons, je l’imagine, l’occasion d’en débattre en séance. La commission est en revanche revenue sur l’allocation de fin de contrat. Elle estime que celle ci fait doublon avec les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen (CEC) dont bénéficie tout volontaire effectuant une mission de six mois minimum. Afin de tenir compte de la spécificité du service civique et des volontaires, qui sont très souvent des étudiants ou des jeunes en reprise d’études, nous avons étendu au paiement des frais d’inscription en formation initiale les droits acquis dans le CEC au titre du service civique. Autre point important, le texte ouvre la voie à une aide financière renforcée pour la structure d’accueil en fonction du diplôme, de l’origine ou encore d’une situation de handicap du volontaire accueilli. C’est une forme d’encouragement des structures à choisir des jeunes au profil plus atypique. C’est également dans cette optique que le texte initial prévoyait de porter à 30 ans l’âge plafond pour effectuer un service civique. Cette disposition a fait débat lors de nos travaux en commission. Pour maintenir l’équilibre fragile entre politique en faveur de l’engagement et outil d’insertion professionnelle, j’ai proposé à la commission de porter l’âge limite à 27 ans, soit deux ans de plus que l’âge actuel. Je suis certaine que le débat se poursuivra tout à l’heure lors de l’examen des articles ! Les auteurs du texte souhaitent également renforcer la formation des jeunes volontaires. La commission a inséré une disposition afin que ces formations soient réalisées par un organisme accrédité spécifiquement pour cela. Elle a aussi porté à trois le nombre de jours de formation obligatoire. Le texte ouvre également la voie à tous les organismes agréés pour faire de l’intermédiation. Cette possibilité, qui permet à une structure de porter juridiquement le service civique et de mettre à disposition le volontaire au profit d’une autre structure, souvent plus petite, est actuellement réservée aux associations. Avec ce texte, une intercommunalité pourra par exemple prendre en charge un service civique au profit des communes ou des associations de son territoire. Cette mesure est de nature à faciliter le développement du service civique auprès de petites structures et dans les territoires ruraux. Le texte vise ensuite à mieux valoriser le service civique. Au nom du principe d’égal accès aux emplois publics, la commission a substitué à la prise en compte d’un service civique dans les épreuves d’admissibilité des concours externes une possibilité pour les statuts particuliers de permettre aux anciens volontaires de bénéficier d’une dérogation aux conditions de diplôme ou de titre pour s’inscrire à ces concours. Pour le troisième concours, elle a remplacé la création d’une voie spécifique pour les anciens volontaires par une prise en compte de la durée du service civique dans le calcul de la durée d’expérience professionnelle exigée. Le service civique est ainsi pris en compte de la même manière que les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Enfin, nous avons inclus la durée du service civique dans les périodes pouvant être prises en compte dans le cadre d’une procédure de validation des acquis de l’expérience. Chers collègues, depuis sa création en 2010, le service civique a su montrer toute sa pertinence et se forger une place à part entière auprès des jeunes. Quinze ans après sa création, et alors que notre jeunesse a soif d’engagement, ce texte représente, une nouvelle fois sur l’initiative du Sénat, une étape supplémentaire dans le développement du service civique.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs,

et c’est essentiel. Il y a plus de jeunes en situation de handicap, parce que nous les avons formés et parce que l’Agence du service civique s’engage au quotidien. Le dispositif n’est pas encore suffisamment connu

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quatre mois après l’examen de notre proposition de loi pour une allocation universelle d’études, je me réjouis de voir, une nouvelle fois, le sujet de la jeunesse au cœur de nos débats. En même temps, je dois bien vous l’avouer, je suis relativement perplexe face à ce texte. Oui, le service civique est un marqueur fort des politiques de jeunesse. Alliant la solidarité et l’intérêt général, il s’inscrit dans une volonté d’ouverture et de découverte du monde associatif. Il représente, pour beaucoup de volontaires, un premier pas dans le monde du travail, ainsi que de nouvelles perspectives pour des jeunes en décrochage scolaire ou rencontrant des difficultés pour déterminer leur projet de vie. nous sommes bien clairs : nous sommes pour le service civique ! Mais c’est bien parce que nous sommes pour ce dispositif que nous refusons de fermer les yeux et de faire comme si les contours étaient parfaits et que la seule chose à faire Élargir un tel dispositif sans l’encadrer, c’est prendre le risque de le dénaturer et, surtout, de précariser les premiers concernés, c’est à dire les jeunes. En effet, nous pensons que la montée en puissance du dispositif sur cette dernière décennie ne doit pas nous conduire à une course en avant des chiffres, à vouloir toujours plus de personnes engagées, sans se préoccuper de leur situation, de leur indemnisation et de leur insertion dans le monde du travail. Mes chers collègues, il est de notre responsabilité de repérer, de comprendre et, surtout, de répondre aux limites du service civique.

le retour en arrière en commission sur le niveau d’augmentation de l’indemnité, qui, finalement, n’est pas à la hauteur des attentes. Ces élargissements, sans renforcer les garde fous face au risque d’emploi dissimulé, ne sont pas souhaitables. Dans ce cas, le risque est de voir se développer un service civique à deux vitesses, selon la perspective esquissée par l’étude du Centre les jeunes les plus diplômés qui s’engageraient après une période d’activité par goût de l’intérêt général et, de l’autre, les jeunes moins diplômés qui feraient un service civique après une période de chômage pour trouver une opportunité professionnelle et une source de revenus.

Renforçons le service civique existant et améliorons le dispositif, en augmentant nettement l’indemnité, en nous assurant du respect des missions, en encadrant le temps horaire des volontaires et en proposant dix jours de formation.

Il a prospéré sous la présidence Hollande et trouve son prolongement aujourd’hui, avec comme objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale, en offrant la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans

Premièrement, le service civique ne parvient toujours pas à satisfaire l’un des objectifs pour lesquels il a été créé, à savoir renforcer la mixité sociale dans la société. C’est ce que révèle d’ailleurs le dernier rapport de la Cour des comptes, qui fait état d’une dégradation de la mixité sociale. la convergence entre l’engagement volontaire et l’appropriation des notions d’intérêt général et de citoyenneté demeure fragile. Le service civique est plus considéré comme un moyen pour les jeunes d’acquérir de l’expérience et de faciliter l’accès à l’emploi

l’a rappelé M. Kanner dans son intervention liminaire. Le service civique ne doit pas être le moyen de remédier aux difficultés financières des associations ou au manque de moyens dans les services publics. Nous craignons donc que cette disposition aille à rebours des préoccupations de la jeunesse d’aujourd’hui. En effet, avec un taux de chômage des 18 25 ans de 17,4 % en novembre 2023, la France enregistre un taux supérieur à la moyenne européenne.

Shemseddine avait 15 ans. Il est mort jeudi dernier après avoir été tabassé à Viry Châtillon. Deux jours avant, Samara était, elle aussi, frappée à Montpellier, dans mon département. Des jeunes massacrant d’autres jeunes… Qu’avons nous donc raté ? Cette proposition de loi s’inscrit dans ce contexte de violence, de déni de la vie, si précieuse, sur fond de valeurs oubliées ou jamais acquises. Le service militaire unissait les classes sociales et les niveaux d’études dans un objectif de défense de la patrie et du pays. Les différents gouvernements ont senti qu’il fallait renouer avec un sens commun autour de la République après la fin de la conscription nationale en 1997. Le groupe du RDSE s’est toujours engagé pour ces enjeux.

Comme l’a dit hier matin Fabien Roussel à la radio, ces drames d’une violence extrême sont non « plus des faits divers, mais des faits de société ». Il est donc primordial de revoir l’éducation morale et civique et de revenir aux fondamentaux. La citoyenneté, c’est le civisme, la civilité, la solidarité,

considèrent le service civique comme un véritable projet de société qui mérite d’être redynamisé et souhaitent que le dispositif s’étende à plus de jeunes, quels que soient leur origine, leur situation professionnelle ou leurs projets.

actuellement à la notion de citoyenneté d’initiative, car il existe une différence entre être citoyen et se sentir citoyen. De fait, tous les mineurs et les non nationaux sont exclus de la citoyenneté. Difficile dans ce cas de se sentir membre et acteur de la société ; il faudrait se pencher sur ce problème. Nous alertons sur le risque que le service civique pâtisse des récentes annonces de coupes budgétaires

créé en 2010, consiste en un engagement volontaire de six à douze mois, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, ou à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Il permet aux jeunes de s’investir dans une mission d’intérêt général au sein d’une association, d’une collectivité publique ou d’un établissement public. Le service civique est une chance pour la France.

eux une occasion unique d’acquérir de nouvelles compétences et de développer une expérience professionnelle. Ils peuvent ainsi améliorer leur et augmenter leurs chances de trouver un emploi après leur mission. Le service civique permet par ailleurs de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux horizons et de se développer personnellement. Grâce à lui, les jeunes peuvent gagner en confiance, en maturité et en autonomie. Pour la société ensuite, le service civique constitue un outil précieux pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il permet aux jeunes de se mélanger, de s’entraider et de contribuer à une société plus solidaire et plus inclusive. Le service civique permet encore de sensibiliser les jeunes aux valeurs de la République et de les encourager à participer à la vie de la cité. Il est ainsi un outil essentiel pour la promotion de la citoyenneté et de la démocratie. Il permet enfin de répondre aux défis sociaux et environnementaux de notre époque. Les jeunes peuvent ainsi s’engager dans des missions de lutte contre la pauvreté, l’illettrisme ou l’exclusion ou encore pour la protection de l’environnement. Depuis sa création en 2010, ce dispositif a permis à plus de 780 000 jeunes de s’investir dans des domaines aussi variés que l’éducation, l’environnement, la solidarité ou la culture. Nous examinons aujourd’hui un texte qui vise à le rendre plus attractif et accessible à tous les jeunes. Cette proposition de loi est une étape importante pour le développement du service civique. Si elle est adoptée, elle encouragera plus de jeunes à s’engager dans une mission d’intérêt général, tout en améliorant la qualité des missions et l’accompagnement des volontaires. Elle renforcera l’encadrement légal et valorisera l’engagement citoyen.

Si nous comprenons la volonté de Mme la rapporteure, une extension de la tranche d’âge aurait pu être perçue comme un frein à l’accompagnement des jeunes sur le marché du travail. Par ailleurs, l’âge moyen des volontaires étant de 21 ans, il y a fort à parier que cette mesure n’aurait bénéficié qu’à un nombre très limité d’individus. Les volontaires plus âgés désireux de s’investir dans une mission auront toujours la possibilité de remplir des missions d’urgence en dehors de leur contrat. Enfin, l’allocation de fin de contrat a été supprimée, car elle faisait double emploi avec le compte d’engagement citoyen. Le CEC sera désormais utilisé pour financer les frais d’inscription en formation initiale. Le droit à la réintégration dans le cursus de formation est garanti pour les étudiants en césure. La possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur de prendre en compte un engagement de service civique lors d’une inscription en premier cycle a été précisée. En revanche, l’obligation d’intégrer cet engagement parmi les critères d’accès aux filières sélectives a été supprimée. Enfin, la commission a modifié l’article 3, visant à valoriser le service civique dans les concours de la fonction publique. La question de la rémunération du service civique pose question et mérite d’être retravaillée. Si une revalorisation peut être envisagée, celle ci doit se faire en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Il ne nous semble pas opportun de la faire évoluer dans le cadre de l’examen de ce texte. Pour autant, ce qui fonctionne doit être soutenu. C’est la raison pour laquelle la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. Notre groupe fera de même. Il soutiendra les efforts visant à faire connaître ce dispositif précieux pour renforcer la cohésion sociale, développer la citoyenneté et construire une société plus solidaire. La parole

ce n’est point pour inviter les hauts fonctionnaires de Bercy à méditer sur les réalités de nos territoires, c’est pour rappeler à quel point la place que la formation, l’expérience et l’expérimentation occupent depuis des décennies est essentielle dans le parcours nécessaire d’apprentissage du citoyen. Les violences entre jeunes des derniers jours, qui mènent trop souvent à des conséquences dramatiques, montrent plus que jamais notre besoin de « faire nation

J’adresse mes condoléances et tout mon soutien aux parents, à la famille, aux amis, aux élus de Viry Châtillon et aux équipes pédagogiques dans cette épreuve, plus qu’insupportable. Cet acte montre une nouvelle fois – une fois de trop – qu’il est urgent de sortir de cette spirale de la violence. Bien loin d’être naïfs, nous reconnaissons que le service civique est un moyen – non le seul moyen, mais tout de même l’un des moyens – de lutter contre l’engrenage de la violence qui enlise la jeunesse dans notre société. Il est essentiel de définir ou de redéfinir un cadre qui permette à la jeunesse de donner un sens à son engagement citoyen, à la croisée des chemins des droits et des devoirs, au carrefour républicain de l’utilité et des engagements. À cet égard, le service civique est un outil utile. Depuis sa mise en place par le président Nicolas Sarkozy en 2010, il a fait ses preuves, en montant en puissance sous la présidence de François Hollande. Ce dispositif est en effet plébiscité par les jeunes et constitue un véritable levier d’intégration. S’il ne s’agit nullement d’opposer le service civique au service national universel,

Les dispositions proposées sont vectrices d’intégration, d’autonomie, d’accueil et de vivre ensemble. C’est justement ce dont nous avons plus que jamais besoin. En l’espèce,

Cependant, il faut penser à long terme. Les jeunes en situation précaire doivent pouvoir bénéficier du service civique au même titre que les autres. On ne peut pas fermer la porte aux personnes les plus en difficulté, alors même que ce dispositif mène à une meilleure intégration à l’emploi. Il est donc subséquemment utile pour réduire les charges sociales. Dernière avancée, enfin : la valorisation de l’engagement des volontaires

Il permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s’engager, pendant une période de six à douze mois, auprès de structures pouvant relever des secteurs de la culture, du développement international, de l’action humanitaire, de l’éducation, de la protection de l’environnement, de la santé, de la solidarité, du sport ou encore de la citoyenneté européenne. Depuis 2010, plus d’un demi million de jeunes ont pu effectuer une mission de service civique. Actuellement, plus de 85 000 jeunes par an accèdent pour la première fois à ce dispositif, dont le budget s’élève à environ 440 millions d’euros. Le nombre de missions réalisées a quadruplé en dix ans.

Le groupe des Républicains et apparentés, que je représente, souhaite voter pour ce texte, malgré nos réserves initiales. Nous tenons d’ailleurs à remercier Mme la rapporteure, Sylvie Robert, qui par son travail et son écoute exigeante a permis de rapprocher les points de vue. Un accord semble désormais à notre portée, moyennant quelques ajustements, que la discussion à suivre devrait nous permettre d’obtenir. Nous mesurons aussi l’effort consenti par l’auteur, Patrick Kanner, pour parvenir à un texte à l’ambition mesurée certes, mais susceptible de faire avancer la cause de l’engagement de notre jeunesse. Certains diront que les jeunes ne s’investissent plus dans notre société et semblent se désintéresser de la démocratie. Je ne partage pas pleinement cette analyse. Pour ma part, je considère que c’est notre rôle, en tant que parlementaires, de proposer aux jeunes des outils pour évoluer dans la société et devenir des citoyens.

Ce dispositif est d’autant plus intéressant que nous pouvons y observer une surreprésentation des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, ce qui n’est pas le cas, par exemple, du service national universel, qui accueille principalement des jeunes dont les parents appartiennent aux corps en uniforme.

C’est pourquoi cette revalorisation, si elle n’était pas assortie d’un engagement du Gouvernement d’augmenter dans les mêmes proportions la ligne budgétaire correspondant au service civique, se traduirait par une diminution de 17 000 à 20 000 contrats par an.

La proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui permet d’afficher une volonté que nous souhaitons soutenir, celle de renforcer le service civique. Nous savons toutefois d’ores et déjà que le lien établi entre la Nation et la jeunesse devra, immanquablement et dans un avenir proche, être profondément revisité et réinventé.

Le groupe Les Indépendants Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, aider les habitants au sein de la préfecture pour identifier l’interlocuteur ou le service compétent, animer une épicerie solidaire étudiante,

En encourageant nos jeunes à participer au service civique, nous contribuons à forger des citoyens engagés, conscients des enjeux de notre société et prêts à agir pour la construire ensemble. Nous cultivons ainsi un essentiel sentiment d’appartenance et de solidarité. L’engagement permet également à de nombreux jeunes, parfois fermés et perdus, de s’ouvrir et de s’accomplir. du dispositif en 2010, le nombre de volontaires au service civique est en constante progression. En 2023, près de 150 000 jeunes ont contribué activement à faciliter et à améliorer leur quotidien et celui des autres. C’est une année record. Si le service civique a fait ses preuves, son développement est conditionné à des efforts pour mieux faire connaître, reconnaître et valoriser cette forme d’engagement.

mieux le reconnaître et le valoriser, le texte contient plusieurs avancées auxquelles nous souscrivons. Je pense notamment à la mesure visant à proposer une meilleure formation et à faciliter le parcours étudiant Le texte permet également aux anciens volontaires de participer au paiement de leurs frais scolaires en utilisant les droits acquis au cours de leur service civique. Ce sont des mesures pertinentes.

Pour finir, madame la ministre, je tiens à saluer la création d’un service civique écologique. Je reprends vos mots : « Nous nous sommes attachés à déterminer quelle jeunesse nous voulions laisser à la planète. Nous voulons choisir quelle planète nous allons laisser à la jeunesse.

pour la qualité de son travail, sa précision, mais également pour la qualité de nos négociations. Aujourd’hui, nous nous apprêtons à écrire un nouveau chapitre de cette histoire réussie, ce qui témoigne de l’engouement, de l’efficacité et de la notoriété grandissante de ce dispositif.

Cette démarche pragmatique nous permettra d’évaluer les effets de cette mesure, avant, éventuellement, de la généraliser : il convient de nous assurer que le report de l’âge limite sert véritablement les intérêts de nos jeunes et du dispositif lui même. Il est essentiel que le service civique demeure une expérience enrichissante et accessible pour tous les jeunes, sans que sa qualité ou ses objectifs fondamentaux soient compromis. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les enjeux liés à l’information et à l’accès du dispositif. La proposition de loi vise justement à faciliter cet accès, par le biais du renforcement de l’information auprès des jeunes et de la diversification des missions proposées. Il est crucial que le service civique continue de représenter une opportunité de mixité sociale et d’ouverture, en accueillant des jeunes de tous les horizons, y compris ceux qui sont issus des quartiers prioritaires. Enfin, nous devons veiller à ce que l’engagement des volontaires soit pleinement reconnu et valorisé, dans leur parcours tant éducatif que professionnel. La suppression de l’obligation de prendre en compte le service civique dans les filières sélectives de l’enseignement supérieur et les modifications apportées à sa valorisation dans les concours de la fonction publique

condition d’offrir aux jeunes des missions significatives, encadrées par un tutorat compétent et complétées par une formation civique et citoyenne, que le dispositif pourra pleinement remplir sa mission d’engagement et de cohésion sociale. Il est donc impératif que l’Agence du service civique et les structures d’accueil travaillent de concert pour garantir que les missions proposées répondent aux aspirations des jeunes. Le renforcement de l’information est une autre pierre angulaire de cette proposition de loi. La méconnaissance du dispositif par les jeunes constitue un obstacle majeur à son développement. une campagne d’information ciblée et efficace pour démythifier le service civique, en soulignant sa distinction par rapport à d’autres formes d’engagement ou d’insertion professionnelle, et en mettant en avant son rôle dans la construction d’un parcours citoyen et professionnel. La création d’un cadre juridique pour la participation à des missions d’urgence est une mesure positive : la flexibilité et la réactivité du service civique face aux besoins sociétaux Mes chers collègues, cette proposition de loi nous offre l’occasion de renforcer un dispositif qui a fait ses preuves, en l’adaptant aux défis contemporains. C’est dans une vision de long terme, dans l’esprit de promouvoir les valeurs de citoyenneté et de solidarité, que nous devons aborder les modifications proposées, afin que ce dispositif continue de jouer un rôle clé dans le parcours de vie de la jeunesse. Le groupe Union Centriste est profondément attaché au fait que le service civique reste un vecteur d’engagement citoyen

Le service civique n’a pas échappé à son examen minutieux. Le succès de ce dispositif n’est plus à démontrer : il correspond à une aspiration des jeunes, qui y trouvent un moyen de découvrir ou d’approfondir un engagement citoyen.

mes chers collègues, quelques points de divergence, mais l’essentiel est de renforcer la consistance et la visibilité de ce service civique, sans dénaturer ses missions ni l’éloigner de ses principes fondateurs. La parole

sa pertinence. L’alinéa 7 vise à permettre aux personnes accueillies en France au titre de la protection temporaire de postuler à un service civique. Cette disposition a été ajoutée en commission, sur l’initiative de la rapporteure. Le service civique est déjà ouvert aux personnes de nationalité française, ressortissants des pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers sous certaines conditions, par exemple s’ils justifient d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an.

Madame Billon,

Selon les dispositions actuelles, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser quarante huit heures réparties au maximum sur six jours pour les personnes de plus de 18 ans. Seuls les mineurs âgés de 16 à 18 ans ont une durée hebdomadaire qui ne peut dépasser trente cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours. Le service civique a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et d’encourager l’engagement pour l’intérêt général. Il ne doit pas être utilisé par des organismes pour surexploiter les volontaires, notamment en alourdissant le poids des missions et du temps de travail. Il est essentiel de prévenir de potentielles dérives. Le service civique

Quel est l’avis de la commission ?

l’avis de la commission

quand allez vous prendre conscience de la précarité croissante des jeunes et réagir aux files interminables devant les distributions alimentaires en fin d’année ? Lorsque je me suis rendue à l’une d’elles,

nous nous serions laissé faire, nous aurions apporté un plein soutien à cette proposition et je suis persuadé que Cédric Vial et Stéphane Piednoir auraient retiré leurs amendements. Ce que nous ne voulons pas,

pour s’inscrire aux concours de la fonction publique. Actuellement, cette dérogation est de droit pour les parents d’au moins trois enfants et possible pour les sportifs de haut niveau. Les épreuves et le concours en lui même restent inchangés pour les candidats. Le service civique, d’une durée d’un an maximum – sa durée moyenne est de huit mois –, n’a pas vocation à remplacer des années d’études et par conséquent les titres et diplômes reçus. Le service civique n’est pas un frein à la poursuite des études supérieures ni à la formation et il

que l’accès égal aux emplois publics est maintenu. Il me semble intéressant de valoriser le service civique au sein de la fonction publique. En outre, le droit autorise déjà des dérogations de diplômes et de titres pour les parents de trois enfants et les sportifs de haut niveau. Pourquoi les perchistes qui passent

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.